Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Pouvoirs publics » regroupe les crédits consacrés aux différents pouvoirs publics constitutionnels, à savoir la Présidence de la République, le Parlement, avec l’Assemblée nationale et le Sénat, les chaînes parlementaires, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la République. Elle est régie, je le rappelle, par un principe d’autonomie financière, corollaire du principe de séparation des pouvoirs, selon lequel chaque institution fixe elle même les crédits nécessaires à son bon fonctionnement.

à +1,3 %, les dépenses de fonctionnement, en hausse ces dernières années, le seront de nouveau en 2025, de 11,8 %. C’est particulièrement le cas des dépenses rattachées à l’action présidentielle. Quant aux déplacements de la Présidence, en hausse également depuis plusieurs années, ils affichent néanmoins pour 2025 une baisse de 5 %, soit 20 millions d’euros. Enfin, les dépenses d’investissement

35,25 millions d’euros seraient dévolus aux chaînes parlementaires. L’Assemblée nationale prévoit ainsi pour 2025 un total de dépenses de 643,2 millions d’euros.

il se répartit entre des dépenses de fonctionnement, qui s’élèvent à 366,08 millions d’euros, en hausse modérée de 1,66 %, et des dépenses d’investissement de 12,87 millions d’euros, en augmentation de 2,57 % par rapport à 2024. Au total, en incluant la dotation du Conseil constitutionnel, 16,85 millions d’euros, et celle de la Cour de justice de la République, 984 000 euros, le montant de la mission atteindrait 1,136 milliard d’euros après renoncement aux hausses de dotation, contre 1,156 million d’euros prévus initialement, soit une économie de 20 millions d’euros. La différence, bien sûr, ne va pas résorber le déficit de l’État. Elle est symbolique sur l’exercice. Cet effort n’est d’ailleurs pas nouveau, la dotation étant loin d’avoir été indexée sur l’évolution des prix ces dernières années. Pour ma part, je veux souligner la difficulté sur une longue période de la gestion des pouvoirs publics, avec, en définitive, une absence d’évolution linéaire. On assiste à une forme de compétition,

confrontées à une baisse de leurs fonds de réserve et à des charges importantes pour l’entretien de leur patrimoine historique, les institutions vont devoir disposer de budgets d’investissement importants dans les prochaines années. Cet investissement sera aussi indispensable à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par les pouvoirs publics Je saluais l’année dernière les plans mis en œuvre pour réduire l’empreinte carbone des institutions, mais je m’interroge cette année sur leur soutenabilité, compte tenu des décisions financières prises et des trajectoires fixées pour l’échéance 2050

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient de vous présenter, au nom de la commission des finances, la mission « Conseil et contrôle de l’État et contrôle de l’État », qui rassemble les crédits des juridictions administratives et financières, ainsi que du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Le projet de loi de finances pour 2025 déposé en octobre dernier prévoyait une hausse modérée de 1,8 % des crédits de paiement de la mission pour atteindre la somme modeste de 899,7 millions d’euros. Nous examinerons tout à l’heure un amendement du Gouvernement visant à baisser ces crédits de plus de 7 millions d’euros.

Je m’attarderai tout d’abord sur les crédits de la Cour des comptes et des juridictions financières, qui s’élèvent à près de 261 millions d’euros, en hausse de 2,2 % par rapport à 2024. Les magistrats financiers devraient bénéficier cette année d’une mesure de revalorisation indemnitaire, pour laquelle une enveloppe de 5 millions d’euros est prévue dans le PLF. Cette mesure me semble bienvenue et permettra d’éviter un décrochage de leur rémunération par rapport à celle des administrateurs de l’État. Il serait en effet illogique que les juridictions financières soient confrontées à une perte d’attractivité et paient les conséquences de la réforme de la fonction publique, qui résulte d’une décision gouvernementale. Je salue par ailleurs les efforts de la Cour pour réduire ses dépenses de fonctionnement courant, comme en témoigne la baisse de 5 % des dépenses hors titre 2 du programme. J’en viens maintenant au budget du Cese, qui s’élève à près de 35 millions d’euros, en baisse de 22,4 % par rapport à 2024. Cette diminution des crédits doit toutefois être nuancée, dans la mesure où elle résulte principalement d’une mesure de périmètre. Lors de l’examen du PLF pour 2024, j’avais fait part à notre assemblée de mes réserves sur la budgétisation de l’enveloppe consacrée à la participation citoyenne.

Je conclurai mon propos en évoquant le budget du Conseil d’État et des juridictions administratives, qui concentre à lui seul deux tiers des crédits de la mission. Il s’élève à 604 millions d’euros, en hausse de 3,5 % par rapport à l’année 2024. Cette augmentation des crédits est en grande partie imputable à la poursuite du mouvement de revalorisation indemnitaire des magistrats administratifs, pour laquelle une enveloppe de 8,8 millions d’euros est prévue. L’année 2025 sera par ailleurs marquée par une stabilisation des effectifs des juridictions administratives. Monsieur le ministre, ce gel des effectifs risque de mettre les juridictions administratives sous tension et pourrait conduire à un allongement des délais de jugement.

Je conçois que la stabilisation des effectifs puisse se justifier cette année par la nécessité de redresser nos finances publiques à court terme. Toutefois, la représentation nationale ne pourra pas faire l’économie, lors des prochaines programmations budgétaires, d’une réflexion sur les moyens accordés aux juridictions administratives,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Direction de l’action du Gouvernement », qui réunit les services du Premier ministre ainsi que plusieurs autorités administratives indépendantes telle qu’elle nous est présentée pour 2025, une baisse notable de ses dépenses en crédits de paiement (CP) à périmètre constant. En effet, si ces crédits affichent une légère hausse apparente de 1,23 % à périmètre courant, pour atteindre 1,066 milliard d’euros, cette évolution doit être corrigée de plusieurs transferts en base qui influent sur le périmètre de la mission. À périmètre inchangé, la mission présente une baisse en CP de 14,8 millions d’euros, représentant –1,4 % en euros courants et –3,1 % en euros constants, après correction de l’inflation, pour s’élever à 1,038

2,3 % en euros courants et de 4,0 % en euros constants, le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », qui regroupe les services du Premier ministre à proprement parler, supporte globalement l’ensemble de l’effort budgétaire, passant sous la barre des 900 millions d’euros à périmètre constant.

en euros courants et de 2,6 % en euros constants, pour atteindre un niveau de plus de 140 millions d’euros à périmètre constant. Cette évolution contrastée se retrouve dans les schémas d’emplois des deux programmes. Alors que les efforts de maîtrise des dépenses sur le programme 129 se matérialisent par la suppression de 20 équivalents temps plein (ETP) en 2025, le solde du schéma d’emplois du programme 308 demeure positif, avec 18 ETP supplémentaires en 2025. Au total, le solde du schéma d’emplois de la mission est légèrement négatif en 2025,

ETP. Fort des enseignements de mon récent rapport de contrôle sur le Haut Commissariat au Plan (HCP), je voudrais évoquer la réorganisation des instances de conseil et d’évaluation qui a été engagée par le précédent gouvernement. Ah ! En effet, Michel Barnier avait annoncé la prochaine fusion du HCP et de France Stratégie. M. le ministre pourra sans doute nous préciser l’état d’avancement des travaux sur ce sujet. Pour mémoire, dans le cadre de mon rapport de contrôle, j’avais appelé à la clarification de la répartition des compétences entre le HCP, France Stratégie et le Secrétariat général à la planification écologique. La fusion du HCP et de France Stratégie va plus loin plus loin que ma recommandation initiale. Cette mesure de regroupement peut avoir une valeur d’exemple pour d’autres regroupements de structures administratives, même si les économies budgétaires associées devraient être limitées.

le répète, il me semble que la gestion de ces autorités pourrait être sensiblement améliorée et rationalisée, en particulier dans le domaine immobilier. Aussi, afin d’assurer une contribution des AAI d’assurer une contribution des AAI concernées à l’effort de redressement des finances publiques, la commission des finances propose, par un premier amendement, de geler, à périmètre constant, au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2024 la dotation globale des autorités rattachées au programme 308 Protection des droits et libertés ». Dans le même esprit, la commission propose, par un second amendement, de geler symboliquement la dotation de l’ordre national de la Légion d’honneur. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative administrative ». Géré par la direction de l’information légale et administrative (Dila), celui ci devrait atteindre en 2025 un pic ponctuel de recettes, à 181 millions d’euros, soit une hausse de 8,19 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. Ainsi, alors que les dépenses du budget annexe devraient s’élever à 150,6 millions d’euros en CP, en légère baisse par rapport à 2024, celui ci devrait dégager en 2025 un excédent important, à 30,4 millions d’euros, soit le double du niveau de 2024. Si la Dila prévoit de poursuivre le déploiement des actions de modernisation numérique, la modération des dépenses de personnel pourrait être fortement affectée par une évolution du statut juridique des agents. En effet, le Conseil d’État a remis en cause le statut de de droit privé des agents issus de l’ancienne direction des journaux officiels, qualifiant l’ensemble du personnel d’agents de droit public. Pour conclure, la commission des finances vous propose d’adopter les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » et du budget annexe « Publications officielles et information administrative », tels que modifiés par ses amendements et ceux du Gouvernement. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient depuis maintenant huit ans de vous présenter le budget du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », consacré plus particulièrement à la cybersécurité, la lutte contre les ingérences numériques étrangères et l’appui aux services de renseignement. cyberattaques, la guerre informationnelle, les opérations de déstabilisation des outre mer, ainsi que les tensions causées par les conflits en Ukraine et au Moyen Orient sont reliées à trois sources principales : la Chine, la Russie et l’écosystème cybercriminel.

Ils ont préparé et protégé avec succès les grands rendez vous de l’année 2024 : les élections européennes, puis législatives et, bien sûr, les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)

C’est un outil majeur destiné à l’ensemble des Français, particuliers comme entreprises. Maintenant, qu’en est il pour 2025 ? Avec 425 millions d’euros au lieu de 438 millions, les crédits de paiement de l’action n° 02 « Coordination de la sécurité et de la défense » subiront en 2025 une baisse de 3 % par rapport à 2024. nationale (SGDSN), principalement l’Anssi et Viginum, vont devoir fonctionner avec 8 millions d’euros en moins. Je relève aussi une réduction de 4 millions d’euros des fonds spéciaux et de 1 million d’euros des moyens du groupement interministériel de contrôle (GIC), qui met en œuvre des techniques de renseignement pour les services. nationale (IHEDN), la subvention à ce centre de formation baisse de 3 %, soit 300 000 euros. Pour les effectifs, le plafond d’emplois passe de 1 283 équivalents temps plein travaillé en 2024 à 1 300 pour 2025. Ce budget se caractérise donc par une baisse modeste des crédits et une progression à la marge des effectifs.

À titre personnel, je n’ai pas souhaité entrer dans une logique de transfert de crédits, car il s’agit avant tout d’une responsabilité du Gouvernement. Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen des amendements, d’entre eux plaident pour une hausse des crédits, tandis que le Gouvernement propose, par un nouvel amendement, une baisse de 40 millions d’euros des crédits du programme 129. Les résultats et la motivation des équipes que nous avons rencontrées, avec mon collègue Mickaël Vallet, permettent de penser que la France dispose d’une capacité de premier niveau pour s’adapter et relever les défis.

Les attaques à but lucratif par rançongiciel ont augmenté de 30 % par rapport à l’année passée. Les cibles sont également de plus en plus diversifiées. Par exemple, le secteur du social est de plus en plus visé et devient une source d’inquiétude. Ce secteur ne devra pas être négligé dans le cadre du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, que le Sénat examinera bientôt. Le niveau de maturité des universités et des hôpitaux à cet égard demeure très bas.

L’Anssi va devoir remettre à plus tard plusieurs projets : le passage à l’échelle de l’agence pour mettre en œuvre la directive NIS 2 () devra être retardé ; la création d’un laboratoire dédié à l’intelligence artificielle, qui n’est pas un petit sujet, et d’un second centre de données sécurisé devra être repoussée. Pour la première fois depuis sa création en 2021, le budget de Viginum ainsi que ses effectifs n’augmenteraient pas. Une telle stagnation nous paraît inquiétante, alors que les manipulations de l’information continuent de croître, comme l’a mis en évidence le rapport de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères, présenté

il est aussi incohérent avec les priorités fixées à notre sécurité et à notre défense nationale. C’est pourquoi la commission des affaires étrangères, contrairement aux années précédentes, a donné un avis défavorable

Présidence de la République et la Cour de justice de la République. Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la mission diffère substantiellement de ce qui avait été proposé en 2024, puisque la Présidence de la République ainsi que les présidences du Sénat et de l’Assemblée nationale ont renoncé à leurs demandes initiales.

Les dotations sollicitées par les institutions qu’elle concerne étaient pourtant déjà structurellement insuffisantes pour couvrir leurs dépenses. Au cours des exercices passés, elles ont équilibré leur budget par des prélèvements sur leurs réserves respectives,

à la même date en 2023, elles sont tombées à 3 millions d’euros. Si l’on peut s’interroger sur les moyens humains substantiels qui sont donnés à la Présidence de la République, notamment quand on les compare à ceux des institutions parlementaires, je salue néanmoins sa participation, comme celle des assemblées parlementaires, à l’effort commun qui a été demandé aux citoyens et aux administrations pour le redressement de nos finances publiques. J’attire toutefois votre attention sur une constante, à savoir l’attrition continue des ressources de la démocratie parlementaire. Cet amenuisement des moyens des assemblées pèse sur la capacité d’action des parlementaires. En effet, celle ci dépend en grande partie des moyens humains dont ils disposent pour mener à bien leurs travaux de législation et de contrôle. Or leurs équipes de collaborateurs sont notoirement insuffisantes et ces derniers sont, à notre goût, trop peu rémunérés. J’appelle tout simplement à ne pas refuser le coût de la démocratie parlementaire, essentielle à un fonctionnement équilibré de notre régime politique, notamment pour contrebalancer les moyens d’expertise de l’exécutif. À cet égard, je partage tout à fait les réflexions engagées par mon collègue Grégory Blanc, rapporteur spécial de la commission des finances, qui visent à comparer les moyens alloués

Monsieur le président, monsieur le ministre,

qui a donné des résultats satisfaisants et démontré leur capacité d’évolution. En témoignent la division par deux du délai de publication des travaux d’examen de la gestion, la mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics,

malgré sa diversité, contribue, quoique de manière contrastée, à l’effort budgétaire national. Les crédits de la mission subissent ainsi une baisse de 14,8 millions d’euros à périmètre constant, soit une diminution de 1,4 % en euros courants et de 3,1 % en euros constants, après prise

la régulation des plateformes numériques devient un enjeu crucial à la suite de l’entrée en vigueur du paquet législatif européen relatif aux services numériques. D’autre part, la coordination de la politique numérique de l’État s’intensifie, avec la mise en œuvre de la feuille de route de la direction interministérielle du numérique. occasion, à souligner le rôle stratégique de l’intelligence artificielle, dont les outils en cours de déploiement offrent des perspectives significatives de compétitivité et de productivité dans tous les secteurs de l’économie comme dans les services publics.

internationale. Cet élan doit impérativement être poursuivi et amplifié pour éviter un décrochage et des retards en la matière. Enfin,

Face à ce programme relativement dense, je veux saluer les travaux et la clarté des présentations de nos rapporteurs. Même si tous les sujets abordés méritent d’être débattus, je souhaiterais m’attarder en particulier sur la mission « Pouvoirs publics », qui comprend notamment le budget de la Présidence de la République, ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que celui du Conseil constitutionnel.

Il est donc tout à fait évident que l’augmentation des crédits de cette mission aurait été difficile à justifier auprès de nos compatriotes, d’autant que le Gouvernement ne cesse de déposer de nouveaux amendements d’annulation de crédits, parfois massifs, sur certaines missions essentielles. Je tiens donc à saluer la décision de la Présidence de la République, de notre président Gérard Larcher et de la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun Pivet de refuser l’augmentation des dotations initialement prévue pour cette année. certains postes de dépense posent question et mériteraient davantage de transparence ; je pense notamment aux dépenses liées aux activités présidentielles, dont les frais de réception. Certains de nos collègues auront plus d’ambition puisqu’ils proposeront une réduction supplémentaire de ces budgets. Je pense en particulier à l’amendement que défendra mon collègue Henri Cabanel tout à l’heure. Même si je n’y suis pas favorable, car la démocratie – en particulier une démocratie de qualité – a forcément un coût, je comprends cette position. Elle marque une prise de conscience du sentiment de déconnexion que connaissent nos compatriotes vis à vis de la classe politique. J’aimerais également évoquer le budget du Conseil constitutionnel.

La Cour constitutionnelle italienne dispose ainsi d’un budget de 65 millions d’euros, avec 44 greffiers et 222 agents au total. Le Tribunal constitutionnel espagnol compte 210 agents, pour un budget de 28 millions d’euros. Le Conseil constitutionnel français affiche de son côté un personnel de 87 ETP, en excluant les neuf membres du Conseil. Nous sommes donc loin de nos voisins européens, alors même que le Conseil se transforme peu à peu en véritable cour constitutionnelle, en particulier depuis la mise en place de la Il faudra donc, à un moment donné, que le Conseil puisse bénéficier de moyens en adéquation avec l’importance de ses missions, en particulier pour favoriser la qualité de ses décisions. concerne les deux chambres parlementaires, comme l’a souligné le rapporteur spécial, le refus annoncé des hausses de dotations pour cette année va accroître les déficits de ces institutions, risque de poser des difficultés pour le financement des dépenses, surtout en matière d’entretien du patrimoine historique, patrimoine historique, et aura un impact important sur les fonds de réserve de ces institutions. Mais j’irai plus loin : doter le Parlement de moyens, c’est le mettre en mesure de jouer pleinement son rôle de contre pouvoir face à l’exécutif. C’est lui permettre d’assurer ses missions constitutionnelles sans les brader. Or l’attrition continue des ressources du Parlement pèse sur la capacité d’action des députés et des sénateurs. Oui, nos compatriotes attendent que leurs représentants et les élus soient exemplaires, surtout en matière de dépense publique. Mais les Français veulent aussi une législation de bonne qualité. Ils attendent des parlementaires qu’ils puissent contrôler et évaluer efficacement l’action du Gouvernement.

Alors que les deux chambres du Parlement ont annoncé dès l’automne dernier, par la voix de leurs présidents et de questeurs, un effort notable de participation à la réduction de la dépense publique, il nous faut souligner l’insuffisance des conditions dans lesquelles nous exerçons nos missions constitutionnelles. Ainsi, dans cet hémicycle, nous examinions hier les crédits de la mission « Action extérieure de l’État

nos travaux presque par surprise, là où nous nous étions arrêtés, mais avec des protagonistes différents, des agrégats qui ont changé et des amendements gouvernementaux qui changent la donne à la dernière minute.

Le rapporteur pour avis appelle enfin à « ne pas refuser le coût de la démocratie parlementaire, essentiel à un fonctionnement équilibré de notre régime politique, notamment pour contrebalancer les moyens d’expertise de l’exécutif

ne le fait pas. Cela conduit à donner droit à l’usager, qui est ainsi incité à contester de nouveau. Dépassée, la juridiction administrative avait souhaité que le législateur rétablisse, en l’encadrant, l’obligation d’acquitter le FPS avant de pouvoir le contester. En l’absence d’interconnexion des fichiers, cela pose néanmoins la question de la capacité à rembourser les usagers qui gagneraient leur recours. Sur ce point, mes auditions m’avaient permis de comprendre que, trop souvent, le Trésor public ne serait pas en mesure d’y procéder simplement, notamment parce que les collectivités délèguent le recouvrement des

Chacun sait l’importance des travaux du HCE, aujourd’hui présidé par l’ancienne ministre Bérangère Couillard, qui a remplacé à ce poste Sylvie Pierre Brossolette, dont je salue le travail et l’engagement.

mais je n’ai pas pu trouver par qui, pourquoi ni à quel niveau. Cet exemple dit beaucoup de l’opacité des documents auxquels nous avons accès. En tout état de cause, les travaux du HCE nous sont précieux et je suis favorable à ce que ses moyens soient au moins clarifiés et sanctuarisés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

tous ordres prennent place dans le débat politico médiatique pour cracher leur haine des autres, des femmes, des homosexuels, des étrangers… Il nous faut retrouver – ici, au Parlement – une confrontation saine des idées par le débat démocratique. Or le débat démocratique, cela

Vogel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui des crédits alloués au fonctionnement des institutions de la République. Alors que le Gouvernement acte une baisse nette des dotations de la Présidence de la République ; alors qu’un amendement de nos questeurs acte la baisse des dotations du Sénat, de l’Assemblée nationale et de Public Sénat ; alors que le

Gouvernement persiste, d’investir dans l’avenir que représente la transition écologique, dans l’adaptation à la crise climatique, nous condamne à subir des coûts individuels et collectifs beaucoup plus importants dans les années à venir ; alors que nous discutons, dis je, d’un budget qui se trompe d’économies,

Ces crédits ne sont pas un coût pour le Parlement européen : il s’agit d’une ressource précieuse ! Ils rendent possible l’embauche d’équipes solides, assez nombreuses, expérimentées, correctement rémunérées. Ils permettent d’attirer les meilleurs au service du plus important : la fabrique de la loi, le contrôle de l’exécutif, la démocratie parlementaire, l’intérêt général. Ils rendent le Parlement européen plus fort, mieux à même de bâtir une expertise et une position de négociation indépendantes vis à vis de la Commission et du Conseil. Bref, ils servent la démocratie. Tant que nous persisterons dans le choix de sous doter ce qui nous rend forts, nous resterons un Parlement structurellement faible. Je ne saurais m’y résoudre ! Sans compter que ces déficits de moyens engendrent d’autres coûts.

baisse des réserves, en faisant la course à celui qui coupera le plus dans le fonctionnement des pouvoirs publics, on mettra toujours à mal le pouvoir et le public ! C’est encore la même chose pour Public Sénat. Franchement, à l’heure où Donald Trump vient de prendre le pouvoir aux États Unis, où Elon Musk fait un salut nazi,

qu’il faut renforcer et non menacer. Oui, la démocratie parlementaire a indéniablement un coût, mais ce coût est infiniment faible par rapport à celui de son absence. Réduire les moyens du Parlement ou de la Présidence de la République, réduire les moyens des pouvoirs publics, ne nous économisera rien. Oui, nous devons

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois missions budgétaires sont conjointement étudiées ce matin : « Pouvoirs publics », « Conseil et contrôle de l’État » et « Direction de l’action du Gouvernement

Cette augmentation profitait à toutes les institutions de la mission, à l’exception du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Elle correspondait en partie à une indexation sur l’inflation de la dotation sollicitée. Il a été rappelé que la Présidence de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat ont ensuite annoncé renoncer à la réévaluation qu’ils avaient demandée. Comme ces institutions représentent plus de 95 % des crédits de cette mission, la dotation pour 2025 est en fin de compte globalement constante par rapport à 2024. Il faut évidemment saluer la participation de l’exécutif à l’effort collectif de redressement des comptes publics, même si certaines dépenses nous interpellent encore, en particulier pour les déplacements à l’étranger du Président de la République.

Quant à la démocratie parlementaire, s’il faut admettre qu’elle a un coût légitime, nous approuvons là aussi, contrairement à d’autres, le choix, proposé en conscience et en responsabilité, de renoncer aux augmentations de dotations demandées. Sous ces quelques réserves, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur des crédits

1,83 %, pour atteindre 899,7 millions d’euros. Cette augmentation s’explique notamment par une hausse des dépenses de personnel au sein des juridictions financières. Elle est la bienvenue, particulièrement au regard de la conjoncture économique et financière de la France, dont les déficits avaient été, rappelons le, massivement sous évalués au printemps dernier. Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, le point d’alerte de cette mission réside plutôt dans le fonctionnement insatisfaisant de certaines instances administratives. si le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » voit ses crédits de paiement augmenter de plus de 3 % par rapport à la loi de finances pour 2024, force est – hélas ! – de constater que nombre de ressorts sont encore engorgés et fonctionnent au ralenti, faute de moyens adéquats.

nous appelle à faire montre de vigilance, mais ne nous empêchera pas de voter les crédits de cette mission. Il en sera autrement pour la mission « Direction de l’action du Gouvernement ». Avec ses deux programmes, « Coordination du travail gouvernemental » et « Protection des droits et libertés », cette mission occupe une place centrale dans notre architecture budgétaire, puisqu’elle traduit en actes les priorités stratégiques et organisationnelles de l’État.

dans le contexte de cybermenaces croissantes et d’ingérences étrangères toujours plus fortes, il aurait été opportun de sanctuariser les moyens qui leur sont dévolus, y compris pour les aider à faire face aux nouvelles missions qui leur ont été confiées par de récents textes européens et nationaux.

mais aussi la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, la Défenseure des droits et la Cnil. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’apprête à voter contre les crédits alloués à la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

d’une grande diversité, sont toutes indispensables au bon fonctionnement de notre État de droit. Les différents collègues qui m’ont précédé ont rappelé avec force et une certaine constance notre attachement à ces crédits. de quatre minutes – je m’efforcerai de m’y tenir –, je formulerai juste quelques observations. En premier lieu, la mission « Pouvoirs publics » réunit les crédits de la Présidence

toute augmentation, alors même que la dotation du Sénat est stable depuis de très nombreuses années. Je tiens donc à saluer les efforts du Sénat particulièrement et à rappeler, comme certains de mes prédécesseurs l’ont fait, que cela ne sera pas sans difficulté pour les missions et les programmes du Sénat. Cependant, le rétablissement de nos finances publiques est un effort de tous les instants auquel les acteurs publics doivent contribuer. En agissant de la sorte, le Sénat fait preuve d’une exemplarité dont il faut se féliciter.

Les différentes dotations des trois programmes de cette mission n’évoluent pas de façon identique. Les programmes 164 et 165, qui financent l’activité des juridictions financières et administratives, connaissent une hausse modérée, justifiée notamment par la revalorisation indemnitaire des magistrats administratifs due à la réforme de la haute fonction publique de l’État. Je souhaite à cet égard mettre en avant le travail des juges administratifs et des greffiers,

En dernier lieu, la mission « Direction de l’action du Gouvernement » regroupe des entités très hétérogènes, comme des autorités administratives indépendantes ou des secrétariats généraux, dont le point commun est leur rattachement au Premier ministre. Cette mission connaît, à périmètre constant, une baisse notable des dépenses en crédits de paiement. Je relèverai

République et Territoires promeut des efforts budgétaires dans les ministères et chez les opérateurs qui le peuvent, il a toujours soutenu que l’État doit impérativement tenir ses engagements régaliens. Nous soutiendrons donc les amendements visant à rétablir les modestes budgets de ces opérateurs stratégiques pour notre souveraineté nationale.

nous entamons l’examen groupé de trois missions budgétaires qui ont en commun d’abonder les fonctions centrales de notre appareil d’État : la mission « Pouvoirs publics » pour les crédits de nos principales institutions constitutionnelles, la mission « Conseil et contrôle de l’État » pour les juridictions administratives et financières et la mission « Direction de l’action du Gouvernement » pour la coordination du travail gouvernemental et le fonctionnement de certaines autorités publiques. l’ampleur de ce triple périmètre regroupant un certain nombre de programmes, je ne reviendrai que brièvement sur certains des points saillants de ces différents segments du projet de loi de finances. Tout d’abord, la mission « Pouvoirs publics » présente une singularité : la séparation des pouvoirs conduit à laisser une grande autonomie financière aux institutions qui y sont rattachées, celles ci déterminant elles mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement. il y a lieu de se réjouir que ces institutions aient choisi de participer à l’effort de redressement des comptes publics, en acceptant de renoncer à une hausse de leur dotation pour cette année. Dans ces conditions, les crédits de cette mission s’élèveront à environ 1 137 millions d’euros. Ces crédits, bien qu’ils ne représentent qu’un poste budgétaire somme toute relativement faible, n’en sont pas moins ceux qui alimentent les organes centraux de notre démocratie.

Dans le contexte financier actuel, le Sénat a naturellement aussi fait le choix de renoncer à l’indexation sur l’inflation de la dotation de l’État pour son fonctionnement, d’un commun accord avec l’Assemblée nationale. J’évoquerai aussi brièvement l’une des institutions de la mission, la Cour de justice de la République.

s’élèvera cette année à près de 530 000 euros, contre 497 000 euros l’année précédente, dans le cadre d’un bail courant encore pour plus de six ans. Dans un contexte où de nombreuses institutions judiciaires manquent de moyens et où les fonds alloués aux opérations immobilières d’investissement se raréfient, un effort particulier de bonne gestion immobilière doit être effectué à tous les niveaux.,

tabou. La mission « Conseil et contrôle de l’État » regroupe trois programmes. Ceux ci rassemblent respectivement les moyens alloués au Conseil d’État et au reste de la juridiction administrative, au Conseil économique, social et environnemental, à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. Les crédits de cette mission progressent légèrement, de 1,8 % en crédits de paiement, pour atteindre 899,7 millions d’euros en 2025. Une partie substantielle de cette somme sert à financer les dépenses de personnel du programme 165

La participation de la mission à l’effort budgétaire global est donc largement passée par une stabilisation de la trajectoire des effectifs et une contraction des dépenses hors titre 2. Les efforts déjà importants consentis par les juridictions administratives pour réduire leurs dépenses de fonctionnement du contexte budgétaire et des tendances actuelles sur le terrain, il pourrait malheureusement être compliqué d’atteindre les objectifs en matière de délais de jugement et de baisse du stock des affaires en instance.

de notre ancien collègue François Noël Buffet, et la création des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d’asile permettront de dégager à terme des marges supplémentaires. Enfin, la mission « Direction de l’action du Gouvernement » connaît, elle, une baisse de 3,1 % de ses crédits, après prise en compte des effets de périmètre

la participation des services rattachés au Premier ministre à l’effort de maîtrise des comptes publics, ainsi que la rationalisation de la maquette budgétaire en matière de transformation numérique. En effet, le transfert dans ce programme de la direction interministérielle du numérique figurait à la fois parmi les recommandations de la commission des finances du Sénat et celles de la Cour des comptes. Par contraste, nous observons une dynamique haussière des crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés », qui regroupe de nombreuses autorités administratives indépendantes. Si cette augmentation est souvent le résultat d’évolutions du droit européen, l’attribution de nouvelles missions et le changement de locaux de certaines de ces autorités, telles que la Cnil ou la HATVP, doivent cependant être suivis avec vigilance. À la suite du rapport présenté en 2023 par notre ancienne collègue Nathalie Delattre, les rapporteurs budgétaires ont appelé à un effort de rationalisation du fonctionnement de ces structures

curieuse. Décidément, des marges de manœuvre importantes existent dans ce domaine. Ce volet devra faire l’objet d’une attention particulière lorsque des travaux seront entrepris pour d’autres types de structures publiques, notamment les agences de l’État. Par contraste, félicitons nous au passage de la bonne santé du budget annexe « Publications officielles et information administrative », qui devrait dégager un excédent cette année. C’est là le fruit d’une gestion rigoureuse, qu’il faut saluer, de la direction de l’information légale et administrative, notamment de ses efforts

D’une grande diversité, ces crédits sont tous indispensables au bon fonctionnement de notre État de droit. Ils visent notamment à garantir aux pouvoirs publics, aux organes chargés de leur contrôle, ainsi qu’aux autorités administratives indépendantes qui s’assurent du respect des libertés individuelles les moyens nécessaires à leur action.

Le budget du Conseil constitutionnel sera, lui, réduit d’un million d’euros. J’observe que les six entités de la mission confirment de manière quasi homogène cette constante. Ainsi, et comme l’ensemble des administrations publiques, nous allons travailler à rationaliser nos dépenses. L’objectif sera le même partout : dépenser moins, certes, mais surtout J’en viens à la mission « Conseil et contrôle de l’État ». Les moyens qui lui sont alloués pour l’année 2025 s’inscrivent dans la continuité des orientations stratégiques suivies ces dernières années, notamment dans la programmation du budget 2023 2027 des juridictions administratives. Je me réjouis de l’augmentation de 3,5 % des crédits visant à revaloriser les métiers de magistrat et de greffier. Cela nous permettra de mieux répondre à la progression constante du volume des contentieux, estimée à 5 % en moyenne annuelle depuis près de cinquante Les juridictions financières bénéficieront d’une progression de leur dotation de 2,2 %, corrélée à une activité en hausse. Elle permettra de poursuivre la mise en œuvre de leur feuille de route, notamment « JF 2025 », le projet stratégique des juridictions financières, qui qui a pour objectif de fournir aux citoyens une information plus fiable, de formuler des recommandations plus claires et concrètes pour améliorer les politiques publiques et garantir l’exemplarité de la gestion publique.

dans la mission « Direction de l’action du Gouvernement », je me félicite de la diminution de 12,5 % des dépenses de fonctionnement des cabinets du Premier ministre, des ministres délégués et des secrétaires d’État. De même, je salue l’amendement gouvernemental tendant à prévoir une rationalisation supplémentaire des dépenses de 25,6 millions d’euros relatives aux moyens des administrations relevant du Premier ministre, toujours dans la logique d’exemplarité qui nous honore et nous oblige. Je note les moyens alloués au programme 308 pour renforcer la protection des droits de l’Homme et des libertés publiques et individuelles.

Monsieur le président, madame, messieurs les questeurs, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays a besoin d’un budget. Ce budget nécessite un effort inédit de maîtrise de la dépense publique,

ils visent à garantir aux pouvoirs publics, aux organes chargés de leur contrôle, ainsi qu’aux autorités indépendantes qui veillent au respect des libertés individuelles, les moyens nécessaires à leur action. Ces pouvoirs publics, organes et autorités se doivent, tous, d’être exemplaires, et c’est le cas.

quatre équivalents temps plein lui seront affectés. Cette commission a bénéficié d’un schéma d’emplois positif ces dernières années. Nous pouvons saluer le travail de ce tribunal, à l’image de celui des juridictions administratives et financières.

du Conseil économique, social et environnemental est quant à lui relativement stable, en raison d’une mesure de périmètre, à savoir la pleine mise en œuvre de l’évolution du financement de la caisse de retraite de ses membres, qui n’est plus supporté par le programme 126.

Cette progression résulte essentiellement de la fusion du programme 352 mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du programme 129 « Coordination du programme gouvernemental

Le budget de ce programme augmente ainsi globalement de 4,5 %. Le maintien de cet effort, après plusieurs budgets successifs en progression, traduit bien la volonté du Gouvernement de continuer à accompagner ces autorités dans la croissance de leurs activités et de leurs missions. Je pense en particulier à la Cnil, qui doit prendre en compte le développement de l’intelligence artificielle, à la HATVP, qui est directement concernée par la mise en œuvre de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, et à la Défenseure des droits, dont l’activité connaît une croissance régulière. Les autres Les autres autorités qui ont également bénéficié de la création de postes au cours des dernières années voient leurs moyens reconduits. Pour poursuivre les efforts collectifs de redressement des finances publiques mis en avant par le Gouvernement dans le présent PLF, il vous sera proposé une mesure d’économie, préservant

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la réduction des déficits publics. Le Premier ministre a souhaité que ses services contribuent pleinement à l’effort de l’ensemble des services de l’État.

J’ai évidemment entendu les différents orateurs qui se sont succédé à cette tribune, ainsi que l’inquiétude des rapporteurs et du président Perrin, avec qui nous nous sommes entretenus, sur les besoins croissants de l’Anssi et de Viginum.

Avec des niveaux de crédits qui restent supérieurs à ceux qui étaient prévus dans la LFI 2023, ce budget marque certes un réel effort de réduction des dépenses, mais il ne remet pas en cause la capacité des services à exercer leurs missions. Je le réaffirme : les économies qui vous seront proposées ne mettront pas en cause la capacité des services concernés à exercer leurs missions. C’est ainsi que nous entendons concilier la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et la poursuite, dans de bonnes conditions, de l’action d’intérêt général portée par ces organismes. cet égard, je tiens à remercier MM. les rapporteurs, qui ont produit une étude précise et de qualité des crédits qu’il vous incombe d’examiner aujourd’hui, ainsi que MM. les rapporteurs Cadic et Masset pour le temps qu’ils ont bien voulu m’accorder et pour la pertinence de leurs propositions.

Vous l’aurez compris, sur ces missions budgétaires, comme sur toutes les autres, il sera demandé à la représentation nationale de consentir aux efforts collectifs dictés, non pas seulement par le Gouvernement, mais par les réalités économiques et financières auxquelles nous devons faire face. Je sais pouvoir compter sur la qualité des débats et des travaux du Sénat, même dans les conditions particulières que j’ai rappelées au début de mon propos, pour arriver à un compromis au service du pays et des Français. Mes chers

Monsieur le ministre, en cohérence avec la dotation qui lui a été allouée en application de la loi spéciale du 20 décembre 2024. Au moment où le Gouvernement essaie de maîtriser les dépenses publiques, cet amendement –

Cigolotti. Le Parlement doit participer au redressement des finances publiques que commande l’aggravation des déficits. Le 15 octobre dernier, d’un commun accord, l’Assemblée nationale et le Sénat

qu’il sollicite les questeurs du Sénat afin que ceux ci déposent un amendement de réduction de sa dotation. Le présent amendement, cosigné par les trois questeurs, exauce ce vœu et confirme l’engagement du Parlement en traduisant, dans le PLF, le renoncement à la revalorisation de 1,7 % des dotations des deux chambres la dotation de l’Assemblée nationale serait ainsi réduite de 10 330 009 euros et celle du Sénat de 6 009 000 euros. Par ailleurs, cet amendement tend à réduire les crédits de la chaîne « Public Sénat » de 307 000 euros

à celle d’une étude indépendante faite par nos assemblées, fondées sur le travail des fonctionnaires et collaborateurs, qui occupent aujourd’hui une place grandissante dans l’exercice de notre mandat.

capacité de contrôle. Revenir sur ces crédits, c’est dévaloriser le rôle de l’ensemble de ces institutions. Enfin, on ne peut pas dire qu’il n’est pas possible de baisser

Est ce acceptable ? Je ne le crois pas, sachant que nous partions d’une situation où ils étaient déjà globalement sous payés par rapport à leur niveau d’étude et à leur charge de travail et en comparaison avec les autres pays européens. Par ailleurs, je ne comprends pas l’argument de la droite :

explication de vote.

Monsieur le ministre,

pour mieux rendre compte des nouvelles missions des juridictions financières résultant du plan « JF 2025 », lancé en 2021 par le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il n’est pas question ici de remettre en cause le bien fondé ni le bilan de ce plan, que nous estimons être une réussite. Au contraire, nous souhaitons mettre pleinement en lumière le travail qui a été accompli ces dernières années.

œuvre : depuis 2022, seules quatre saisines ont été effectuées par des collectivités territoriales et les CRC ne se sont saisies elles mêmes que d’une demi douzaine de projets d’évaluation. Nous proposons donc, par cet amendement, de compléter l’objectif « Assister les pouvoirs publics » par un second indicateur qui retracerait l’activité des CRC liée à leur mission d’évaluation des politiques publiques et d’avis sur les projets d’investissement exceptionnels. Contrairement à l’indicateur « Nombre d’auditions au Parlement il s’agirait là d’un indicateur que la Cour des comptes pourrait partiellement maîtriser, puisque les chambres régionales peuvent s’autosaisir. Ce nouvel indicateur permettrait ainsi de ne pas limiter au seul Parlement le suivi dans le projet annuel de performance de la fonction d’assistance aux pouvoirs publics effectuée par les juridictions et d’en favoriser une lecture davantage territorialisée.